Quel est l'avis du Gouvernement ?

comme l'a affirmé le Gouvernement le 9 septembre dernier devant l'Association française pour l'hydrogène et les piles à combustible. La stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène doit pouvoir être déclinée sur le territoire à l'échelon régional de la même manière que l'on entend dans le présent texte décliner le développement des énergies renouvelables. Il ne saurait y avoir de découplage territorial entre les deux stratégies. Quel est l'avis de la commission ? Nous ne pouvons que partager l'intention des auteurs de cet amendement. J'émets cependant deux réserves. La première, c'est que l'amendement vise l'énergie hydrogène ; or, d'un point de vue rédactionnel, il me semble plus pertinent de faire référence à l'hydrogène bas-carbone. La deuxième, c'est que je me demande s'il est réellement pertinent de prévoir d'ores et déjà une répartition régionale des capacités de production d'hydrogène

Malhuret. Cet amendement vise à associer les collectivités territoriales d'une même région à la définition des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables. Ce préalable ne peut concourir qu'à la réussite des politiques à conduire puisque ces collectivités seront ensuite invitées à suivre les indicateurs et la méthodologie retenue pour le déploiement et la mise en oeuvre de ces objectifs régionaux. Quel est l'avis de la commission ?

L'avis est favorable.

minimaux pouvant être dépassés. Le Conseil d'État, dans son avis sur le présent projet de loi, n'a pas manqué de relever que le rapport de compatibilité n'empêche absolument pas une région de retenir dans son Sraddet des objectifs supérieurs sont fixés dans le décret. Il convient de noter d'ailleurs que les Sraddet pris dans leur ensemble conduisent pour certaines filières à des objectifs de développement des énergies renouvelables bien supérieurs à ceux qui sont identifiés dans la PPE. Pour ces différentes raisons, le présent amendement vise à préciser ce point de manière claire et sans ambiguïté.

En effet, face à l'urgence climatique, nous devons soutenir le développement des EnR comme le solaire, le gaz renouvelable, la géothermie, l'hydroélectricité, mais de manière planifiée, comme nous l'avons déjà souligné

? Comme l'a rappelé le Conseil d'État dans son avis, on peut déjà déduire du texte que les régions pourront fixer des objectifs supérieurs aux objectifs régionaux prévus par décret. J'entends néanmoins la préoccupation des régions qui souhaitent poursuivre une politique ambitieuse de développement des énergies renouvelables. La précision rédactionnelle que tendent à introduire ces amendements identiques me semble satisfaisante. J'émets donc un avis favorable. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Cet amendement vise à préciser l'implication des autorités en charge des PCAET dans les stratégies régionales de promotion des énergies renouvelables. En effet, la promotion des énergies renouvelables dans les territoires doit prendre appui sur les PCAET, qui se généralisent peu à peu sur l'ensemble du territoire national. Ils constituent le cadre de territorialisation des objectifs nationaux et régionaux de nos politiques énergétiques et climatiques. C'est pourquoi, dans un souci de cohérence et de coordination des différents échelons territoriaux, il semble fondamental d'impliquer très étroitement les autorités chargées de ces documents dans la définition des stratégies régionales. Quel est l'avis de la commission ? La commission estime que cet amendement complète utilement les travaux menés au sein de la commission, qui ont permis d'assurer une meilleure association du bloc communal au comité régional des énergies renouvelables. L'avis est donc favorable. Quel est

destiné à être le lieu privilégié d'information et de consultation des collectivités territoriales et des citoyens de la région sur les questions ayant trait à l'énergie. Ce comité sera en particulier chargé de proposer

très concrètement avec les régions de la stratégie économique de déploiement des énergies renouvelables. Quel est l'avis de la commission ? Les contrats de plan État-région ont vocation à financer les projets exerçant un effet levier pour l'investissement local, dont la transition écologique et énergétique. Cet amendement tendant à préciser que ces contrats contribuent à l'atteinte des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables me semble donc le bienvenu. L'avis est favorable.

aux enjeux de transition énergétique et climatique. Ce volet, à hauteur de près de 4,6 milliards d'euros de crédits d'État, est l'un des premiers en termes financiers, vous le savez.

Cet amendement vise à ce que la déclinaison régionale des objectifs nationaux de développement éolien soit cohérente avec la superficie et le potentiel de production des territoires favorables à l'implantation d'éoliennes. l'organisation par le préfet de région d'un recensement sur l'ensemble du territoire régional des zones susceptibles d'accepter l'accueil d'éoliennes, par une consultation des élus. Les réponses données à cette consultation auraient une valeur contraignante puisqu'il ne serait plus possible d'autoriser l'exploitation d'éoliennes dans les communes ayant indiqué y être défavorables. En effet, l'impact de ces installations nécessite que leur implantation se fasse avec l'accord des communes concernées ne puisse aboutir malgré l'opposition des habitants et des élus du territoire d'implantation, comme c'est le cas actuellement. L'avis favorable d'un territoire n'exonérerait ainsi pas un projet d'implantation d'éoliennes des procédures d'autorisation existantes. Le dispositif proposé complète ainsi utilement l'amendement de notre collègue Édouard Courtial, qui prévoit une consultation à valeur contraignante des conseils municipaux. Les élus des territoires ayant indiqué lors de la consultation être être favorables à l'accueil d'éoliennes garderaient ainsi la main pour refuser ou accepter un projet d'implantation.

du productible du site d'implantation du projet. Il s'agit de favoriser une répartition aussi équilibrée que possible des installations sur l'ensemble du territoire et de faciliter l'atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Une telle mesure me semble importante.

M. Martin Lévrier. Dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, puis de la loi relative à l'énergie et au climat, la France s'est fixé un objectif d'au moins 40 % d'énergies renouvelables dans sa production électrique la réalisation de tels projets peut constituer une gêne pour les installations et équipements de nos armées. Afin de permettre la réalisation des projets éoliens, qui contribuent à la transition énergétique, notre défense est entrée dans une logique partenariale avec les industriels qui exploitent ces parcs par le biais de conventions prévoyant le financement d'équipements permettant de pallier cette gêne. Mais, à la suite d'une ordonnance du 26 janvier 2017, l'autorisation environnementale unique a remplacé toutes les autorisations auxquelles ces projets étaient soumis. Cela a entraîné de fait la dispense de permis de construire pour les projets de construction d'éoliennes soumis à autorisation environnementale. Sans remettre en cause l'autorisation environnementale unique, il apparaît donc nécessaire de prévoir un dispositif similaire à celui qui était en place, afin de rendre applicable ce système collaboratif entre nos armées et nos parcs éoliens. Quel

qui permettait de couvrir les moyens supplémentaires de sécurité aérienne induits par l'installation d'éoliennes, est devenu inapplicable en 2017 Pourquoi la question n'a-t-elle pas été anticipée dans la rédaction de l'ordonnance de 2017, qui a instauré des dispenses de permis de construire ? Deuxièmement, le problème des interférences entre les éoliennes et les radars aériens est connu depuis près de vingt ans. À l'heure où nous cherchons à développer les énergies renouvelables, quel est

des collectivités, protection des consommateurs, prix unique de l'électricité et propriété publique des réseaux. Au-delà de ces modifications, elle a voulu conforter l'objectif de décarbonation du texte en comblant plusieurs lacunes sur l'hydroélectricité, notre première source d'énergie renouvelable, sur le nucléaire, au fondement des trois quarts de notre mix énergétique, ainsi que sur l'hydrogène renouvelable et bas-carbone, énergie largement évoquée mais peu soutenue. À cette fin, elle a repris les dispositions de la proposition de loi tendant à inscrire l'hydroélectricité au coeur de la transition énergétique et de la relance économique, adoptée par le Sénat le 13 avril dernier. Elle a aussi fixé le principe selon lequel aucun réacteur nucléaire ne peut être arrêté en l'absence de capacité équivalente de production renouvelable nouvelle. Enfin, elle a introduit pour l'hydrogène un cadre stratégique et des mécanismes incitatifs. Ce serait une première législative

à des appels d'offres pour favoriser le développement des capacités de stockage d'électricité en vue de répondre aux besoins de flexibilité du système électrique. Le gestionnaire de réseau serait ainsi tenu de conclure des contrats avec des lauréats des appels d'offres pour leur apporter un soutien financier selon les modalités prévues dans ce cadre. L'amendement vise à compléter le dispositif en permettant que le gestionnaire de réseau de transport soit compensé des charges qu'il supporte en application de ces contrats des charges de service public de l'énergie. Cela existe déjà pour d'autres dispositifs de soutien en matière d'électricité.

tellement gros qu'on ne le voit plus. Madame la ministre, vous le savez mieux que personne, on aura beau bricoler tout ce qu'on voudra, interdire les vols sur les trajets courts, passer au Oui Pub, réemployer les bouteilles, bref contraindre chaque instant de la vie des Français, on ne parviendra pas à la neutralité carbone sans le nucléaire ! C'est pourquoi il nous semblait impensable que le présent projet de loi, colonne vertébrale de la stratégie française de la transition climatique, reste muet sur le sujet. Nous nous sommes donc félicités de l'introduction de l'article 22 BA. Néanmoins, le texte est largement perfectible. Il énonce que les fermetures de réacteurs nucléaires prévues par la loi Énergie-climat ne peuvent être décidées

comprendre que les capacités renouvelables actuellement constituées autorisent la fermeture de x réacteurs ? Cette imprécision majeure est d'ailleurs relevée par le Gouvernement dans l'exposé des motifs de son amendement de suppression.

Le dispositif proposé n'a donc, en l'état actuel, aucune chance de ralentir le rythme de fermeture des réacteurs, puisque la production de l'ensemble des énergies renouvelables actuellement disponibles en France représente 30

souligne l'importance de ce terme -de production d'énergies renouvelables permettant de fournir un volume d'énergie équivalent à la production des réacteurs nucléaires dont la fermeture est programmée.

à la mise en service de capacités de production d'énergies renouvelables permettant de produire un volume d'énergie équivalent à celui provenant des réacteurs nucléaires dont la fermeture est programmée.

de s'assurer que les actions de maîtrise des consommations d'électricité et de déploiement des capacités de production d'électricité renouvelable ont bien été engagées à un niveau suffisant pour permettre la fermeture de ces centrales sans compromettre l'équilibre du système électrique. Bref, on ne s'interdit plus d'avancer, à condition de le faire dans le

tout arrêt de réacteur nucléaire doit s'accompagner de la mise en service de capacités de production d'énergies renouvelables équivalentes. Ces arrêts ne sauraient en effet conduire à accroître la production et la consommation d'énergies fossiles, bien souvent importées. Il est donc urgent de conforter notre sécurité et notre souveraineté énergétiques, en veillant à ne pas déstabiliser davantage notre système électrique par des arrêts de réacteurs nucléaires mal calibrés, car mal évalués.

À ce stade, je souhaiterais rappeler la robustesse de notre sûreté nucléaire, qui s'articule autour de deux établissements complémentaires, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), chargé d'une mission

Si les projections faites aujourd'hui dans le cadre de la prochaine

sans exclusive dans la lutte contre les dérèglements climatiques, dès lors qu'elles ne sont que très faiblement émettrices de gaz à effet de serre, la décarbonation de notre modèle étant notre objectif.

préciser que la production d'énergie de substitution à l'arrêt de réacteurs nucléaires doit être effective, continue et pilotable. Ce sont des précisions intéressantes permettant de garantir

Je voudrais remercier le groupe Union Centriste de cette précision qui tend à consolider notre sécurité d'approvisionnement- c'est important pour nos concitoyens et pour notre économie. Cette mention vient conforter l'intention initiale de la commission dont l'amendement tend à la mise en service de telles capacités. La commission des affaires économiques n'a pas pu prendre

la programmation pluriannuelle de l'énergie, le Gouvernement a en réalité fragilisé notre souveraineté énergétique et même confronté notre pays à un risque de ruptures régulières de son approvisionnement électrique. son approvisionnement électrique. RTE a bien identifié cette situation qui nécessite, il faut le rappeler, de relancer régulièrement nos centrales à charbon, fortement émettrices de CO2, et d'importer une énergie dont, par définition, on ne maîtrise pas le coût.

sur lequel tout le monde, me semble-t-il, peut s'accorder et qui est conforme aux attentes des Français : aucune fermeture de réacteur nucléaire ne peut intervenir sans l'assurance de capacités de production d'énergies renouvelables équivalentes.

de notre mix énergétique met nécessairement nos capacités de production sous tension. Je rappelle que nous sortons d'un hiver au cours duquel RTE a placé notre pays en situation de vigilance particulière. D'après le gestionnaire, cette situation doit perdurer jusqu'en 2023

et compensée par un effort d'innovation et de recherche sur le nucléaire du futur. Il s'agit de reprendre le leadership que notre pays exerce depuis les années 1960 sur un secteur industriel fondamental, qui est gage de notre souveraineté énergétique et de la sûreté d'approvisionnement pour tous les Français.

un garant de l'empreinte carbone faible du mix électrique français- c'est une évidence ! L'objectif de remplacer les énergies fossiles pour répondre à nos objectifs climatiques est bien sûr nécessaire et urgent, nous le savons tous ici. D'ailleurs, madame la ministre, sans remettre une pièce dans le juke-box du débat sur les éoliennes et sans nuire à votre densité capillaire, je partage votre analyse sur la stérilité d'un débat manichéen du pour ou contre l'utilisation, vieille comme le monde, de l'énergie du vent. Ce que j'ai dit hier soir de façon un peu vive, et je m'en excuse, c'est que son nécessaire développement dans le bouquet énergétique, pour reprendre l'expression de mon ami Jean-Louis Borloo, doit être compris et accepté par les populations locales avec l'aval des conseils municipaux. Il me paraissait important de faire cette précision. Les énergies renouvelables peuvent à l'évidence aider à atteindre nos objectifs, mais sans remplacer pour autant et pour l'instant l'énergie nucléaire. dernière présente l'avantage d'être bon marché, pilotable, c'est-à-dire en capacité de produire de l'électricité de manière prévisible, et surtout mobilisable à tout moment. Compte tenu de l'électrification massive de notre économie, en particulier dans le secteur

En effet, le nucléaire en tant qu'énergie décarbonée est un garant de l'empreinte carbone faible du mix électrique français. L'objectif premier est de remplacer les énergies fossiles pour répondre à nos objectifs climatiques. Les énergies renouvelables peuvent contribuer à cet objectif, mais elles ne peuvent pas remplacer l'industrie nucléaire qui a l'avantage d'être bon marché et pilotable. Une réduction trop rapide de notre parc nucléaire par la fermeture de réacteurs pourrait créer un effet contraire et déstabiliser le réseau électrique. Ce scénario de 55 % de nucléaire et de 45 % d'énergies renouvelables en 2035 est le scénario dit Volt du bilan prévisionnel de 2017 de RTE. Il permet la réduction la plus rapide et importante des émissions

vous proposez d'interdire que le volume d'électricité cédé à un fournisseur au titre de l'Arenh puisse alimenter un consommateur pour la part de son offre de fourniture d'électricité couverte par des garanties d'origine renouvelable.

Toutefois, l'Arenh est lié au fournisseur d'électricité qui choisit ou non d'exercer son droit d'accès à l'électricité nucléaire historique. Il n'est en revanche pas possible de tracer la part d'électricité Arenh dans une offre de fourniture donnée. Ainsi, le mécanisme que vous proposez serait difficile à mettre en oeuvre en pratique. De plus, il ne répondrait pas à son objectif : un fournisseur pourrait s'y conformer sans changer ses approvisionnements, en affectant arbitrairement ses volumes d'Arenh à la partie non couverte par des garanties d'origine renouvelable de ses offres commerciales. Considérant que le mécanisme proposé ne serait pas opérationnel et que le futur label de l'Ademe permet de répondre au besoin de transparence vis-à-vis du consommateur sur l'Arenh, j'émets un avis défavorable.

6,5 gigawatts de capacité d'électrolyse doivent être installés à l'horizon 2030, et nous avons un objectif de production de 600 kilotonnes d'hydrogène décarboné, pour une consommation qui est aujourd'hui de 900

qui opposait les pro-éoliens, qui seraient anti-nucléaires, et les pro-nucléaires, qui seraient des anti-éoliens. Je crois que c'est un peu plus complexe que cela. Je vais d'ailleurs le démontrer, puisque cet amendement s'inscrit s'inscrit dans le prolongement de ce que vient d'exposer Ronan Dantec sur l'hydrogène produit à partir d'électrolyse et d'énergies renouvelables, en l'occurrence des éoliennes. Cet amendement vise à créer une nouvelle dérogation légale pour autoriser les raccordements indirects d'installations de production d'hydrogène à très faibles émissions de gaz à effet de serre, tout en conservant, pour les consommateurs qui le souhaitent, la possibilité d'exercer leurs droits comme s'ils étaient raccordés au réseau de distribution publique, par l'installation d'un dispositif de décompte géré par le gestionnaire du réseau public de distribution. Cela permettra d'accélérer le déploiement et la croissance de la production Je citerai l'exemple d'une unité de production qui est en cours de construction en Vendée, à partir d'éoliennes installées dans le secteur de Bouin. Quel est l'avis de la commission

dans nos territoires. Avant d'envisager une telle modification, il est préférable de s'assurer de l'absence d'incidence juridique ou financière négative. C'est pourquoi je demande l'avis du Gouvernement. Quel est l'avis du Gouvernement ?

rien n'empêche un producteur d'avoir une installation d'électrolyse associée à son installation de production. En revanche, dès lors qu'il s'agit de deux installations distinctes, le réseau public est, et doit rester, le moyen de raccordement privilégié. Il n'y a aucune raison qui nous semble justifier une dérogation pour ce type d'installation. Cette disposition remettrait directement en cause le réseau public d'électricité en permettant des installations de consommation non raccordées au réseau public. c'est sur lui que pèsent les obligations de qualité et de desserte. Un raccordement entre consommateur et producteur n'offrirait aucune garantie au consommateur, notamment en cas de problème, par exemple sur l'installation électrique du producteur. L'électrolyseur n'aurait alors plus aucune garantie de pouvoir consommer de l'électricité depuis le réseau. Je le répète, il n'est pas souhaitable d'introduire une dérogation générale pour un type d'utilisation. S'agissant de la traçabilité de l'origine renouvelable de l'électricité, ce n'est pas le lien direct entre les deux installations qui la garantit. D'une part, l'électrolyseur consommera à des moments où des EnR ne produiront pas et, d'autre part, à certains moments, l'électrolyseur ne consommera pas ce qui est produit. La question de l'origine renouvelable continuera donc de se poser. Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à votre amendement. Quel est donc l'avis de la commission des affaires

Cet amendement vise à permettre aux régions, départements, communes et à la Ville de Paris de participer activement au développement de la filière de l'hydrogène décarboné, tant pour utiliser l'hydrogène comme carburant pour le transport public que pour décarboner l'industrie, en partenariat avec des industriels. Il s'agit d'une clarification juridique nécessaire pour accompagner l'émergence de la nouvelle filière de l'hydrogène. n° 2209 rectifié. Les évolutions proposées dans l'amendement sont intéressantes. Ces modifications, toutes facultatives, sont positives. Elles sont complémentaires du paquet législatif sur l'hydrogène, que la commission des affaires économiques a adopté.

Il s'agit d'un amendement qui vise à créer un régime transitoire pour les concessions hydroélectriques autorisables qui sont échues. Les ouvrages hydroélectriques de moins de 4,5 mégawatts relèvent du régime de l'autorisation, et non de celui de la concession, qui s'applique aux puissances supérieures. Cependant, ce seuil a été relevé au cours du temps. Il existe donc de vieux ouvrages de moins de 4,5 mégawatts qui font l'objet d'une concession, car le seuil était plus bas lors de leur création. Ces ouvrages, qui sont appelés des concessions autorisables, ont vocation à revenir au régime de l'autorisation à la fin de leur concession. Cela nécessite une procédure administrative longue, complexe, pour sortir l'ouvrage du domaine public, puis le mettre en vente avec mise en concurrence. Or, du fait de la longueur de cette procédure, certaines concessions autorisables échues avant 2016 n'ont pas pu être mises en vente avant leur échéance, et se trouvent maintenant dans une situation de vide juridique. L'amendement que je vous présente a pour objet de créer un régime transitoire, avec un cadre juridique clair, qui permettra de finaliser les procédures, tout en ayant la possibilité de prendre des mesures de police environnementale et, pour l'exploitant, de procéder aux travaux qui n'avaient pas pu être réalisés à cause de la situation de vide juridique. Pour éviter de mettre les exploitants face à un mur d'investissements, des dispositions sont prévues, y compris la possibilité de délivrer à l'exploitant une autorisation d'occupation temporaire sans mise en concurrence, d'une durée maximale de sept ans, afin de permettre l'amortissement d'une partie de ses investissements. Cet amendement vise, vous l'aurez compris, à combler un vide juridique qui conduit à bloquer des investissements nécessaires à la remise en bon état des installations et à faciliter leur cession et, partant, la poursuite de leur exploitation, en rassurant notamment le futur exploitant, qui n'aura pas à supporter le coût de travaux non réalisés. Il s'agit donc d'un amendement de simplification pour l'hydroélectricité de taille modeste. Quel est l'avis de la commission

de nous soumettre une évolution aussi substantielle à un stade si avancé du projet de loi, d'autant que cette disposition n'a fait l'objet d'aucune évaluation préalable quant à ses incidences juridiques et financières. Ensuite, le dispositif pourrait entraîner un lourd report de charges de l'État vers l'exploitant de la concession échue.

Or cette énergie bas-carbone et locale est aujourd'hui négligée dans les textes de planification de l'eau. Afin d'inscrire dans le droit le potentiel de la petite hydroélectricité, nous proposons une modification

Les précédentes estimations avaient exclu sans raison 95 % de sites hydroélectriques que l'on peut équiper aujourd'hui. Il importe, mes chers collègues, de remédier à ce non-sens énergétique et économique,

pour les porteurs de projets hydroélectriques. Elle pourrait aussi s'avérer plus contraignante. Le Sénat a d'ores et déjà adopté des dispositifs de soutien très complets à l'hydroélectricité dans le cadre du présent projet de loi. Je demande le retrait de l'amendement, sinon l'avis sera défavorable.

suite d'une concertation avec garant menée par l'État du 19 avril au 30 juin 2019 sur le projet de prolongation de la concession du Rhône, et au regard de la spécificité de cette concession, qui s'étend sur plus d'une dizaine de départements, et de sa triple mission, il

des affaires économiques ? Le présent amendement aurait pour conséquence de substituer l'État au département dans l'exercice d'une compétence relative à l'hydroélectricité. En l'absence de concertation exhaustive des conseils départementaux concernés, il n'est pas souhaitable d'y procéder. Si des évolutions de compétences locales doivent avoir lieu, elles peuvent intervenir dans le cadre du projet de loi 3DS, examiné prochainement par le Sénat. C'est une demande de retrait, sinon l'avis sera défavorable. évidemment un avis favorable sur cet amendement. Les cahiers des charges des concessions hydroélectriques prévoient qu'une partie de l'électricité produite est reversée aux acteurs locaux, en pratique sous la forme d'une compensation financière. cet amendement, il est prévu que, pour la Compagnie nationale du Rhône, la liste des bénéficiaires soit arrêtée par le préfet. Cette particularité est pleinement justifiée par la particularité de la concession du Rhône, dont les ouvrages s'étendent sur plus d'une dizaine de départements, et qui a une triple mission- cela a de production électrique et d'usages agricoles. Aussi, il est nécessaire de préserver une vue d'ensemble sur les usages des énergies réservées de la concession afin d'assurer la cohérence et la bonne réalisation de ces missions. Je mets aux voix l'amendement

L'article 22 C intègre dans le projet de loi les dispositions de nature fiscale de la proposition de loi tendant à inscrire l'hydroélectricité au coeur de la transition énergétique et de la relance économique, que nous avons examinée au début du mois d'avril 2020. nous avons défendue lors de l'examen de cette proposition de loi, nous proposons la suppression de l'article 22 C. Tout en partageant la volonté de développer l'hydroélectricité, et particulièrement la petite hydroélectricité, nous doutons de la pertinence et de l'efficacité de ces exonérations, qui bénéficieront surtout à des installations déjà existantes et fonctionnant bien. Les nombreuses exonérations fiscales proposées se traduiront de surcroît par un abaissement des recettes pour le budget de l'État et des collectivités territoriales. En effet, le caractère facultatif de ces exonérations fiscales pour les collectivités territoriales risque d'avantager les territoires les plus riches au détriment des territoires pour lesquels les ressources fiscales sont essentielles. Un dispositif d'aide, notamment à l'installation des infrastructures, nous apparaît bien plus adapté qu'une accumulation d'exonérations. je vous remercie ailleurs, les allégements fiscaux seront obligatoires, s'il s'agit de l'État, et facultatifs, s'il s'agit des collectivités territoriales. Enfin, je précise que la rédaction retenue est bien celle issue des travaux réalisés des finances du Sénat, Mme Christine Lavarde, qui a permis d'enrichir le texte initial en le rendant plus protecteur encore des deniers publics de nos collectivités territoriales. C'est une demande de retrait, sinon l'avis sera défavorable.

211-1 du code de l'environnement prévoit d'ores et déjà que soit assurée la valorisation de l'eau comme ressource économique, en particulier pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable. Nous avons eu un long débat sur cet hier. Comme le droit en vigueur intègre déjà toutes les formes d'électricité, y compris celle dédiée à l'autoconsommation, l'intérêt d'un article supplémentaire ne nous a pas paru évident.

L'article 22 I, tel qu'il est rédigé, fixe un objectif de 50 gigawatts offshore à l'horizon 2050, alors même que l'Ademe estime le potentiel éolien offshore français à 30 gigawatts. Il est important de comprendre les objectifs chiffrés que nous votons : 50 gigawatts, ce sont plus de 90 parcs éoliens offshore supplémentaires, de 70 à 80 mâts chacun 50 gigawatts, ce sont encore de 5 000 à 7 500 éoliennes supplémentaires en mer, ce qui équivaut à tapisser l'intégralité de notre littoral sous prétexte d'écologie.

6,2 gigawatts à l'horizon 2028. Il s'agit de rester sur un rythme concerté et raisonnable de développement de l'éolien offshore. Ce délai permet une réévaluation des objectifs à moyen terme et un engagement progressif et prudent dans cette stratégie qui engage nos côtes.

dont l'objectif, en 2050, est consolidé par le présent article. Tout d'abord, nous prévoyons de veiller à l'accord préalable des communes ou de leurs groupements intéressés dans la mise en oeuvre concrète de cet objectif. En effet, l'information et l'association des élus locaux

territoriale et,, leur acceptabilité sociale. Premier point, une faible visibilité, notamment depuis les communes concernées, afin de préserver la qualité des paysages côtiers, qui constitue un atout précieux pour l'activité touristique des communes littorales. Deuxième point, un faible impact sur les fonds marins ou les activités de pêche en encourageant l'éolien flottant, en sus de l'éolien posé.

dans la mesure où l'éolien en mer constitue l'un des moyens de diversification de notre mix énergétique. Aujourd'hui, on sait tous que la productivité, qui est liée à l'intermittence, est bien plus importante pour l'éolien en mer que pour l'éolien terrestre.

Certes, il peut paraître un peu prématuré d'inscrire dans la loi un objectif de 50 gigawatts à l'horizon 2050, surtout sans discuter des autres objectifs énergétiques à cette date. Encore une fois, je suis attachée aux programmations pluriannuelles, donc je reste cohérente.

ce qui s'est passé lundi à Saint-Brieuc, avec une pollution marine de 170 litres d'huile qui se sont répandus en mer. Néanmoins, pendant ces dix années, nous n'avons pas perdu notre temps, même si l'on peut trouver que c'est long. Il faut savoir que la méthode d'identification des sites, dont on parlait hier, a été éprouvée, et qu'elle est maintenant robuste. Elle se fait par façade maritime, comme Mme la ministre l'a rappelé précédemment, et des zones de moindre contrainte sont identifiées, ce qui conduit à une acceptation et à un consensus sur l'usage partagé de la mer. On a également fluidifié les procédures administratives d'autorisation,

On ne peut donc pas dire aujourd'hui que la concertation n'existe pas : elle est réelle ! La Commission nationale du débat public a rendu son avis, les collectivités de la communauté urbaine de Dunkerque ont pu s'exprimer ; aujourd'hui, tous les feux sont au vert pour que ce projet puisse avancer et garantir l'indépendance énergétique de la France.

d'au moins 70 % des déchets ne pouvant faire l'objet d'une valorisation matière d'ici à 2025, de manière à éviter l'enfouissement de millions de tonnes de déchets. Après avoir extrait de ce gisement toutes les matières recyclables, il restera des refus de tri,

Or seule une faible part des CSR est aujourd'hui valorisée sous forme de chaleur et d'électricité. Il convient donc d'accélérer leur mobilisation, notamment par de nouvelles voies de valorisation, afin d'éviter l'enfouissement des refus de tri. de préciser dans le code de l'environnement que la valorisation énergétique des CSR est également possible dans les installations ayant pour finalité la production d'autres énergies que la chaleur ou l'électricité ; je

Quel est l'avis de la commission sur ces amendements ?

Cependant, comme toute ressource en plein essor, elle présente le risque d'une surexploitation et d'une surconsommation qui viendraient répondre à un marché en pleine expansion et à une demande toujours croissante.

renouvelables. Économiquement, de tels projets peuvent tout à fait contribuer à la relance de l'économie grâce à la création d'une importante activité au niveau local, ainsi que dans toute la chaîne d'approvisionnement, sur laquelle la France est bien positionnée. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement. Il a pour objet, au vu de l'expérience acquise à ce jour, de permettre l'attribution de plus de 1 gigawatt de puissance installée par an d'ici à 2024. Il s'agit d'une évolution nécessaire pour poursuivre l'accélération du déploiement de l'éolien en mer et en tirer tous les bénéfices, que ce soit du point de vue énergétique ou sur le plan économique.

sources de production d'énergie renouvelable : je veux parler des sources houlomotrices ou hydroliennes. En la matière, nous avons la capacité d'assurer la production des outils permettant de générer cette énergie importante pour l'avenir.

Ces technologies ont connu ces deux dernières années une forte accélération. Elles atteignent leur maturité et sont prêtes à être déployées dans des projets pilotes d'envergure. L'établissement de tels objectifs est structurant pour la mise en place d'une planification de long terme. Comme il a été maintes fois rappelé dans cet hémicycle, nous nous devions de développer des énergies renouvelables

ne concerne que les raccordements sur les réseaux de distribution. Si cette disposition était maintenue telle quelle, elle introduirait un biais au dispositif de droit à l'injection et à la cartographie des zonages mis en place par la Commission de régulation de l'énergie, pour retenir la solution de raccordement des installations de biométhane la plus efficiente d'un point de vue technico-économique. La rédaction proposée vise ainsi à augmenter de 40 % à 60 % le plafond de la réfaction des coûts de raccordement aux réseaux de distribution, mais aussi de transport de gaz naturel dont peuvent bénéficier les installations de production de biométhane. Quel civil. Quel est l'avis de la commission dans la mesure où cette disposition a déjà été adoptée par l'Assemblée nationale et par le Sénat, l'évolution proposée par l'amendement mérite d'être examinée avec attention. Je sollicite donc l'avis du Gouvernement. Quel est

pour une durée déterminée et pas nécessairement sur un terrain qu'ils occupent en vertu d'un bail rural. Or la réglementation actuelle, plus particulièrement l'application combinée des articles du code rural qui qualifie l'activité agricole, et L. 411-1, qui qualifie le bail rural, aurait pour conséquence un risque de requalification de ces contrats de location d'unités de méthanisation en baux soumis au statut de fermage. La réglementation actuelle est susceptible de poser de sérieuses difficultés juridiques et opérationnelles pour le développement de nouveaux modèles économiques permettant aux exploitants agricoles de diversifier leurs activités, de valoriser leurs déchets à un moindre coût et à un moindre risque. Il serait opportun de favoriser le renvoi du bail d'unité de méthanisation aux dispositions générales du louage des choses au sein du code civil, afin de ne pas appliquer le régime du fermage. Un modèle locatif permettrait aux exploitants agricoles de ne pas avoir à financer la construction de l'installation, laquelle reposerait ainsi sur le bailleur.

d'unités de méthanisation à destination d'agriculteurs et de faciliter le financement de ce type d'installations, il est nécessaire d'insérer une exception au chapitre I du livre IV du code rural et de la pêche maritime, renvoyant le bail locatif d'unités de méthanisation aux dispositions du code civil. Quel

La France s'est fixé l'objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050, ce qui exige de développer massivement et rapidement la production d'énergies renouvelables en substitution aux énergies fossiles. La production de biogaz est, à ce titre, indispensable pour décarboner certaines activités, notamment industrielles, pour lesquelles la consommation de gaz est difficilement substituable. Une obligation d'incorporation de biogaz dans le gaz vendu par des fournisseurs permettra d'accroître progressivement la part de biogaz livrée aux consommateurs. Cet amendement tend à imposer aux fournisseurs de gaz naturel une obligation de restitution à l'État de certificats de production de biogaz ; les fournisseurs pourront s'acquitter de cette obligation nouvelle, soit en produisant directement du biogaz, soit en acquérant des certificats auprès de producteurs qui ne bénéficient pas d'un soutien par tarifs d'achat. Les producteurs bénéficieront ainsi d'un revenu associé à la commercialisation des certificats de production de biogaz venant s'ajouter aux revenus de la vente physique. Les coûts de la production additionnelle seront ainsi financés par les fournisseurs et les consommateurs de gaz naturel. Ce dispositif de certificats de production de biogaz a été étudié pendant plusieurs mois. Une consultation publique a été menée en février 2021, afin de recueillir l'avis et la critique des acteurs intéressés, et ces travaux ont permis d'intégrer à cet amendement plusieurs améliorations

La prise en compte des certificats de production de biogaz dans les offres de fourniture permettra à l'ensemble des consommateurs de bénéficier d'une part de gaz renouvelable, et l'ajout d'une possibilité d'exonération pour les fournisseurs ayant un faible niveau d'activité permettra de préserver

prévoit, quant à elle, que le biogaz atteigne 7 % de la consommation de gaz en 2030, pourvu que les baisses de coût visées dans la trajectoire de référence, qui sont particulièrement ambitieuses, soient bien réalisées. Toutefois, nous le savons, les contraintes qui pèsent sur les finances publiques contraintes risquent de mettre à mal l'objectif fixé par la loi. cet amendement la mise en place d'un mécanisme de certificats de production, ou CP, de biogaz injecté, reposant sur une obligation de détention de ces CP par les fournisseurs de gaz naturel sur le territoire français, français, qui se les procureraient auprès des producteurs. Dans ce cadre, l'État imposerait aux assujettis de disposer, chaque année, d'un volume de CP proportionnel au volume de gaz naturel livré à leurs clients. Des dispositions spécifiques pourront être prévues pour le gaz naturel livré à des consommateurs industriels, afin de préserver leur compétitivité. Parallèlement, l'État confierait à un organisme indépendant la mission de certifier les installations, de délivrer les CP aux producteurs et de vérifier leur acquisition par les assujettis. Le mécanisme prévoit également des modalités de sanction en cas de non-respect de l'obligation de détention des CP ou de manquement à la réglementation. Comme le prévoit le droit européen, ces CP ne seraient pas liés aux garanties d'origine, afin que ces dernières puissent être commercialisées librement par les producteurs. Enfin, les assujettis auraient la liberté de s'associer au sein de structures communes dédiées ayant pour but de les aider à remplir leur obligation de détention de CP vis-à-vis de l'État. Pour garantir un prix stable et pérenne permettant aux producteurs de prendre les décisions d'investissement et de réduire leur coût de financement, des contrats d'achat à long terme seraient conclus entre ces structures et les producteurs retenus à la suite de procédures de mise en concurrence fondées sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

notamment le gaz verdi. Il est donc proposé un mécanisme de certificats verts, ou CV, reposant sur une obligation de détention de ces certificats par les fournisseurs de gaz naturel sur le territoire français, qui se les procureraient qui se les procureraient auprès des producteurs. Par ce contrat, la structure s'engagerait à verser au producteur de biogaz injecté, pendant une certaine durée, une contrepartie qui est la différence entre le prix garanti remis par le producteur dans le cadre d'un appel d'offres et un prix de référence observé sur le marché. Le producteur recevra cette différence si le prix garanti est supérieur au prix du marché et la reversera dans le cas contraire. La parole est à M.

pour l'alimentation humaine, pour l'alimentation animale, pour les fibres, pour l'énergie, pour la fumure, pour la faune et la flore

collègue. Les dispositions législatives relatives aux missions de service public des opérateurs de l'énergie, notamment des gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel, ne comportent pas de mention de la contribution de ces opérateurs à la recherche des objectifs de neutralité carbone. Or certains gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel peuvent contribuer à ces objectifs et à l'atteinte des objectifs de la PPE, au travers de projets locaux d'efficacité énergétique, auprès d'industriels, voire d'acteurs publics locaux. Afin de permettre à ces gestionnaires de réseaux, acteurs de favoriser l'émergence des projets d'efficacité énergétique, il convient de compléter les missions des gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel transport de gaz naturel mentionnées à l'article L. 111-47 du code de l'énergie. L'émergence de ces projets doit s'inscrire dans le respect du principe d'indépendance

n° 849 rectifié . Il convient de remarquer que les dispositions législatives relatives aux missions de service public des opérateurs de l'énergie, notamment des gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel, ne comportent pas de mention de la contribution de ces opérateurs à la recherche des objectifs de neutralité carbone. Or certains gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel adopté des politiques volontaristes de réduction de leur empreinte carbone, notamment par la mise en place de programmes « éviter, réduire, compenser ». Afin de permettre la reconnaissance pleine et entière de ces programmes à la lutte contre le changement climatique dans le cadre d'une régulation des marchés de l'énergie, il convient de compléter les missions des gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel dans le code de l'énergie. Cet amendement vise à prévoir l'approbation de ce programme par la Commission de régulation de l'énergie, afin que cette dernière puisse évaluer la pertinence technico-économique du programme proposé par le gestionnaire de réseau.

qui concerne l'amendement n° 850 rectifié , l'activité de commercialisation de solutions d'efficacité énergétique est très éloignée de celle de gestion des réseaux de transport de gaz naturel, pourrait créer des problèmes concurrentiels. Je suis donc défavorable à une telle extension du champ d'activité des gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel. Les

ministre. Cet amendement technique vise à préciser les dispositifs de complément de rémunération et de contrat d'expérimentation pour la production de biogaz, afin de permettre leur mise en oeuvre. Quel est l'avis de la commission des affaires

Cet amendement tend ainsi à modifier les modalités de signature des contrats d'achat et de compléments de rémunération de biométhane ; à préciser les modalités de contrôle et de sanction en cas de non-respect de la réglementation et à prévoir l'exercice, par les gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz, d'une mission de comptage du biogaz des installations non raccordées au réseau. L'absence de délai d'application pourrait avoir une incidence lourde sur les contrats pendants ou sur les sanctions encourues. Compte tenu de l'application des remboursements prévus, il est préférable de ne pas adopter ce dispositif, dont les conséquences juridiques et financières sont incertaines.

Il est donc proposé d'augmenter la quantité de chaleur renouvelable devant être produite afin qu'un réseau de distribution de chaleur puisse être classé par une collectivité territoriale. En 2018, la consommation de chaleur distribuée représente 2,4 % de la consommation finale d'énergie. Au cours des trente dernières années, la quantité de chaleur livrée a été multipliée par elle a vocation à augmenter davantage à l'avenir. La décarbonation des réseaux de distribution de chaleur est donc un investissement impératif. La chaleur renouvelable dans les réseaux de distribution de chaleur représente 56 % de la production en 2017. Pourtant, le contenu moyen de CO2 reste élevé, en raison, notamment, de la présence persistante de combustibles à haute teneur en carbone comme le charbon ou le fioul. Le recours accru aux énergies renouvelables pour la production de chaleur est une solution efficace pour réduire l'empreinte carbone des réseaux de distribution et augmenter la part de chaleur renouvelable livrée. C'est pourquoi cet amendement vise à fixer le seuil à 70 %, au lieu de 50 à prévoir que la mesure prendra effet au 1 janvier 2024, afin de laisser le temps aux gestionnaires des réseaux de faire des travaux. Il pourrait être accordé un délai supplémentaire pour les cogénérations gaz, jusqu'à l'échange de leur contrat en cours.

Dans un contexte de forte baisse des prix du gaz, un certain nombre d'industriels saisissent l'occasion et, contre toute logique, basculent en approvisionnement au gaz, prétextant des difficultés d'approvisionnement en bois. bois. Les professionnels de la filière bois sont pourtant formels : ils disposent de grandes quantités de bois, car les déboires des filières papeteries et les volumes sans précédent mis sur le marché du fait des dépérissements sanitaires et climatiques des derniers mois conduisent à un engorgement préjudiciable à toute la filière. Ce qui est aujourd'hui en jeu, c'est tout autant le respect des objectifs de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre que la qualité de la sylviculture menée dans nos forêts et l'approvisionnement des entreprises pour répondre aux objectifs de la Il importe donc de revoir le taux d'approvisionnement en biomasse nécessaire pour bénéficier des avantages fiscaux, afin de le porter de 50 % à 60 %. Tel l'objet de cet amendement. S'il y a effectivement baisse de l'activité de la chaufferie, mesurée par l'Ademe, il pourrait être mis en place, de manière exceptionnelle, des compensations par report de volumes non consommés aux années suivantes, afin de ménager la situation financière des fournisseurs et l'atteinte des objectifs de neutralité carbone. Quel est l'avis de la commission des affaires

En effet, l'approvisionnement des chaufferies en bois peut, s'il est mal géré, menacer le maintien du puits de carbone forestier. Il est important que la stratégie pour la mobilisation de la biomasse forestière respecte une hiérarchie des usages et que le bois utilisé pour la production énergétique provienne en priorité des déchets des coproduits de l'industrie, ou qu'il soit issu de haies gérées durablement. Si la priorité n'est pas donnée à ces ressources au sein de la filière est de voir se développer trop fortement la récolte d'arbres à des fins spécifiques de combustion, ce qui, d'après de nombreuses études, induirait une augmentation trop rapide des émissions de carbone

Des modélisations montrent que pour atteindre les objectifs de neutralité carbone en 2050, il nous faudrait augmenter fortement notre linéaire de haies.

stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévoit déjà des objectifs relatifs à la gestion durable du bois et à l'utilisation des chaufferies au bois. Le bois « durable » ne se limite pas aux déchets ni aux sous-produits de l'industrie du bois.